Le compte rendu intégral de la séance du vendredi 16 novembre 2018 a été publié sur le site internet du Sénat. Il n'y a pas d'observation ? ... Le procès-verbal est adopté. En application de l'article L.O. 319 du code électoral, le mandat sénatorial de M. Jacques Mézard, dont les fonctions gouvernementales ont pris fin le mardi 16 octobre 2018, a repris le samedi 17 novembre 2018, à zéro heure. En conséquence, le mandat sénatorial de Mme Josiane Costes a cessé le vendredi 16 novembre, à minuit. Conformément à l'article 1de l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution, acte est pris de la cessation, le vendredi 16 novembre, à minuit, du mandat sénatorial de M. Didier Guillaume, nommé ministre par décret du 16 octobre 2018 relatif à la composition du Gouvernement. En application de l'article L.O. 320 du code électoral, M. Bernard Buis l'a remplacé en qualité de sénateur de la Drôme. Le mandat de notre collègue a débuté le samedi 17 novembre 2018, à zéro heure.

pour suspicion de fraude fiscale nous montrent à quel point ce sujet est grave et combien les autorités japonaises le prennent au sérieux.

Mes chers collègues, je suis très heureuse de saluer en votre nom la présence, dans notre tribune d'honneur, d'une délégation de l'Assemblée nationale de la République de Bulgarie, conduite par M. Tsvetan Tsvetanov, député et président de la commission parlementaire de la sécurité intérieure. La délégation est accompagnée par Mme Marta de Cidrac et M. Jean-Yves Leconte, tous deux vice-présidents du groupe d'amitié France-Bulgarie, lequel est présidé par notre collègue M. Loïc Hervé, retenu par un voyage d'études à l'étranger. Cette visite s'inscrit dans le cadre du programme de coopération du ministère de l'intérieur avec la Bulgarie. Arrivée ce matin à Paris, la délégation s'est entretenue avec les membres du groupe d'amitié. Elle sera accueillie demain à l'Assemblée nationale, où elle rencontrera plusieurs de nos collègues députés, afin d'échanger sur le thème des politiques de sécurité. Les relations entre la France et la Bulgarie sont anciennes, et les relations interparlementaires contribuent pour une large part à la qualité de notre relation bilatérale. Mes chers collègues, en votre nom à tous, permettez-moi de souhaiter à nos homologues du parlement bulgare la plus cordiale bienvenue au Sénat français, ainsi qu'un agréable et fructueux séjour à Paris. J'informe le Sénat que

J'informe le Sénat que des candidatures ont été publiées pour siéger au sein d'une éventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion sur le projet de loi de finances rectificative pour 2018.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

monsieur le rapporteur général, mesdames, messieurs les sénateurs, j'ai le plaisir de vous présenter le projet de loi de finances rectificative pour l'année 2018, qui s'inscrit dans la démarche de sincérisation de nos comptes publics, engagée par le Gouvernement et par moi-même depuis le début de la mandature. Sincérisation, d'abord, car si le collectif budgétaire n'est plus un exercice de rattrapage de la loi de finances, c'est avant tout parce que la loi de finances initiale pour 2018, dont vous avez eu à discuter, a construit le budget sur des bases assainies.

Le constat est clair : au cours des exercices passés, le collectif budgétaire de fin d'année était devenu une sorte de « voiture-balai »- votre commission des finances, monsieur le rapporteur général, l'a longtemps dénoncé -, emportant avec elle toutes les dispositions n'ayant pas pu être inscrites dans le projet de loi de finances dont l'examen est cependant concomitant.

majorités, la plupart des dispositions figurant dans les derniers collectifs budgétaires, dont la majeure partie était de nature fiscale, n'avaient aucune incidence sur l'équilibre de l'année en cours. C'est pourtant bien le but du projet de loi de finances de fin de gestion

De la même manière, le collectif budgétaire avait vocation à pallier les insuffisances de crédits budgétaires d'une année sur l'autre, notamment dans l'urgence, se contentant de ratifier un décret d'avance qui, cependant, ne nécessitait pas d'autorisation des commissions des finances. Comme je m'y étais moi-même engagé, monsieur le président de la commission des finances, je suis heureux de vous dire que le Gouvernement auquel j'appartiens et le ministre du budget que je suis n'ont présenté aucun décret d'avance pour cette année. Nous terminerons ainsi l'exercice

très nombreux et d'un montant très important, qui ne passaient pas en séance publique. Au cours des derniers exercices, vous l'avez vous-même constaté, le niveau des ouvertures de crédits s'est substantiellement accru,

Nous nous sommes engagés à ce que, dorénavant, les ouvertures de crédits supplémentaires fassent toutes l'objet d'un vote du Parlement, ainsi que de possibles amendements, discutés en séance, sans mesures fiscales, dans le cadre d'une loi de finances spécifique. C'est le cas cette année.

De la même manière, nous ne soumettons aucun décret d'avance à l'avis de votre commission des finances, conformément à l'engagement que j'avais pris devant vous. Si ce PLFR est voté, l'intégralité des ouvertures et des annulations de crédits sur le budget général aura donc été décidée par le Parlement, que ce soit dans le cadre du projet de loi de finances ou du projet de loi de finances

deux articles concernent les ajustements de recettes, qui arrêtent le montant de ressources affectées aux comptes d'affectation spéciale « Transition énergétique » et « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » ; un article technique de ratification de décrets relatifs à la rémunération de services rendus des articles prévoyant, conformément à l'article 11 de la loi de programmation des finances publiques, adoptée l'an dernier sur l'initiative de votre commission, de modifier les plafonds d'emplois des ministères et des budgets annexes, afin de ramener, dès 2018, l'écart entre les plafonds votés par le Parlement et la consommation effective des emplois à un niveau proche de 1 %. Tous les élus locaux le savent, le compte administratif diffère souvent du budget, ce que les chambres régionales des comptes leur reprochent. Aujourd'hui, l'État doit faire l'effort en corrélation, comme vous le demandez, monsieur le rapporteur général, ses effectifs budgétisés et ses effectifs réels. Le texte présenté devant vous suffit à démontrer la prudence des prévisions du Gouvernement, ce que l'on a pu lui reprocher, ainsi que la sincérité des hypothèses retenues. Sincérité s'agissant du cadrage macroéconomique, tout d'abord, puisque la prévision de croissance de 1,7 % pour l'année 2018 reste inchangée par rapport aux hypothèses révisées dans le PLF pour 2019. C'est conforme à la loi de programmation des finances publiques.

Le ratio de dépense publique reste lui aussi inchangé, à 54,6 % du PIB, tout comme le solde structurel, qui s'établit toujours à moins 2,2 % du PIB en 2018. Enfin, l'objectif national d'évolution des dépenses d'assurance maladie, devrait, selon l'avis du comité d'alerte du 15 octobre dernier, être respecté également. Sincérité, enfin, parce que l'évolution des recettes a un effet neutre, si bien que le taux de prélèvements obligatoires s'établit, comme prévu dans le PLF, à 45 % en 2018. La sincérité de notre politique budgétaire, c'est aussi la confirmation du redressement de nos finances publiques. Dans les faits, le solde présenté, révisé à moins 81,3 milliards d'euros dans le PLF 2019, s'établit ainsi à moins 80 milliards d'euros, sous l'effet de plusieurs facteurs dont vous me permettrez d'exposer rapidement le détail. Premièrement, le solde du compte retraçant les participations financières de l'État s'améliore, à hauteur de 1,2 milliard d'euros, grâce à la cession par l'État de 2,35 % du capital de l'entreprise Safran. Deuxièmement, comme nous l'avions annoncé dans le projet de loi de finances pour 2019, notre schéma de fin de gestion nous permettra de dépenser 600 millions d'euros de moins que l'objectif fixé en loi de finances initiale, tout en ouvrant les crédits indispensables au règlement des dépenses obligatoires. Je pense naturellement aux opérations extérieures et intérieures du ministère des armées- 400 millions d'euros -, aux dépassements prévus pour les dépenses de personnel de certains ministères- un T2 qui, notamment à l'éducation nationale, mais également à l'intérieur, représente 300 millions d'euros la prime d'activité- 200 millions d'euros -, pour l'allocation des demandeurs d'asile - 100 millions d'euros -, pour les aides personnelles au logement- 100 millions d'euros -, ainsi que pour les exonérations sur le périmètre de l'outre-mer, pour environ 100 millions d'euros. Ces ouvertures, que chacun pourra qualifier d'urgentes, seront intégralement gagées par des annulations à due concurrence, dans le respect strict du principe de responsabilité des gestionnaires, que nous avons affirmé dans le cadre de la loi de finances initiale pour 2018, et que vous avez soutenu. concernent pour l'essentiel des crédits préalablement mis en réserve, ou bien sont rendues possibles par la réalisation d'économies au-delà de ce qui était initialement prévu. De ce point de vue, les ministères sont responsabilisés. Je vous rappelle que nous sommes passés de 8 % à 3 % de gel,

que, l'an dernier, pris sans doute par les difficultés héritées de la gestion précédente, il m'avait fallu attendre le 27 décembre pour dégeler l'intégralité des crédits, ce qui, convenez-le, n'était respectueux ni de votre autorisation d'engagement ni de la responsabilité des gestionnaires. Voilà, mesdames, messieurs les sénateurs, les lignes directrices de ce collectif budgétaire de fin d'année, qui est conforme aux engagements que nous avons pris devant vous depuis le début de la mandature. Si votre assemblée vote ce texte, prochain, nous permettra, pour la première fois depuis trente ans, et, conformément aux engagements que j'ai pris devant vous, de faire en sorte qu'aucun décret d'avance ne soit déposé par le Gouvernement. Loin de remettre en cause les prérogatives du Parlement, le recours à un PLFR « allégé » est ainsi un instrument de revalorisation de l'autorisation parlementaire, donc du contrôle des membres du Parlement sur les choix budgétaires réalisés.

Certes, l'économie française a retrouvé un peu de dynamisme au troisième trimestre, après un premier semestre très décevant, mais, malheureusement, la reprise est plus faible que nous ministre, votre hypothèse de croissance, fixée à 1,7 %, est peut-être un peu optimiste. Je n'insisterai pas, même s'il est peu probable que l'économie française accélère suffisamment pour permettre d'atteindre ce taux sur l'ensemble de l'année. En tout cas, le rebond nécessaire pour atteindre cet objectif apparaît difficilement compatible avec l'orientation des enquêtes de conjoncture. La consommation des ménages ne semble pas suivre la hausse de leur pouvoir d'achat au dernier trimestre. Nous sommes loin de « l'automne du pouvoir d'achat » que vous prôniez,

L'enquête menée en octobre dernier auprès des chefs d'entreprise dans l'industrie manufacturière fait état d'une baisse de 5 points des prévisions d'investissement pour 2018 par rapport à l'estimation de juillet dernier. D'ailleurs, le Haut Conseil des finances publiques qualifie votre prévision de croissance d'« un peu élevée S'agissant de la trajectoire budgétaire, l'objectif de déficit devrait être tenu, mais c'est un minimum, compte tenu de son manque d'ambition. Le projet de loi de finances rectificative reprend ainsi la prévision de 2,6 % du PIB retenue dans la loi de finances pour 2019,

plus, cette amélioration n'est malheureusement pas imputable à la politique du Gouvernement, puisqu'elle tient à ce que l'on peut appeler la « composante non discrétionnaire » de l'évolution du solde structurel. S'agissant de la situation budgétaire de l'État, le déficit présenté est de 80 milliards d'euros, soit une légère amélioration par rapport à l'estimation initiale de 81,3 milliards d'euros que nous avons examinée la semaine

Le rebasage des plafonds d'emploi au titre de l'année 2018 correspond ainsi à une diminution de 10 805 équivalents temps plein travaillé. Les plafonds d'emplois vont enfin pouvoir être un outil de pilotage des effectifs.

que la question de l'accompagnement de la transition énergétique sera l'objet de toutes nos attentions lors du PLF 2019. Pour notre part, nous contestons le fait que la fiscalité énergétique soit avant tout considérée comme une fiscalité de rendement. Malgré la baisse de presque 600 millions d'euros des « dépenses pilotables », les dépenses sont globalement en hausse de 500 millions d'euros par rapport à la dernière estimation.

compensées par des annulations de crédits des autres programmes de la même mission. Le Gouvernement n'applique donc pas l'article 4 de la loi de programmation militaire, qui pose le principe de solidarité interministérielle

Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, nous ouvrons aujourd'hui la discussion du projet de loi de finances rectificative de l'année en cours, avant de débattre du projet de loi de finances pour l'année à venir. C'est une innovation qui, il faut le dire, est la bienvenue Le schéma de fin de gestion 2018 nous apporte en effet un éclairage utile, avant d'examiner les demandes de crédits de chacune des missions budgétaires pour 2019. Avec le rapporteur général, j'avais plaidé, il y a quelques mois, pour un collectif budgétaire de fin d'année resserré, limité aux seuls mouvements de crédits et mesures fiscales de l'année en cours,

Nos propositions pour renouveler les modalités d'examen des textes budgétaires consistaient à permettre au Parlement de travailler dans de meilleures conditions, moins dictées par l'urgence, afin de connaître réellement l'impact des mesures que l'on lui demande d'adopter.

ministres. Ces modalités d'examen parlementaire ne sont donc acceptables que si le collectif ne modifie pas substantiellement les équilibres de la loi de finances initiale, au risque, sinon, d'affaiblir considérablement la portée de celle-ci et le sens de l'autorisation parlementaire. Par ailleurs, nous constatons que la centaine d'articles que comptait d'habitude le collectif de fin d'année se retrouve littéralement déversée dans le projet de loi de finances. Il s'ensuit un nombre considérable d'amendements de séance, dont certains font plusieurs pages, sans avoir été précédés Nous sommes donc encore très loin d'un progrès des méthodes gouvernementales ! Il faudra, à l'avenir, que ces dizaines de mesures fiscales et budgétaires, ajoutées en cours d'examen parlementaire sur l'initiative ou à l'incitation du Gouvernement, trouvent leur place dans le projet de loi initiale pour être examinées de manière sereine et réfléchie. J'en viens maintenant aux dispositions de ce collectif budgétaire. Il ne modifie pas les hypothèses de croissance économique pour l'année en cours, établies à 1,7 % du produit intérieur brut. Il confirme un déficit public hauteur de 2,6 % du même PIB, soit une toute petite réduction de 0,1 point par rapport à l'an passé. Pour autant, je souhaiterais relever deux aspects qui me paraissent importants au regard des débats qui vont nous occuper sur le projet de loi de finances. Tout l'annulation de 600 millions d'euros de crédits du compte d'affectation spéciale « Transition énergétique ». Avec cette annulation, le produit de la TICPE va alimenter encore davantage le budget de l'État, la fiscalité énergétique servant ainsi à boucler les fins de mois de l'État. Cette économie sera-t-elle consacrée à des objectifs environnementaux ou viendra-t-elle en soutien aux économies d'énergie ? le crédit d'impôt pour la transition énergétique, le CITE, n'ont pas été suivies d'effet. En tout état de cause, l'an prochain, la TICPE financera le budget de l'État à hauteur de 17 milliards d'euros, un record absolu. Le pouvoir d'achat de nos concitoyens s'en ressentira.

Cette annulation sur un budget en baisse augure de nouvelles restrictions l'an prochain, alors même que le marché de l'emploi n'a pas témoigné d'un retournement spectaculaire, c'est le moins que l'on puisse dire. Par ailleurs, ce sont les missions « Recherche et enseignement supérieur et « Écologie, développement et mobilité durable » qui subissent le plus d'annulations dans ce collectif. J'estime que les annulations sur ces thématiques sont autant de signaux négatifs sur les capacités de notre pays à préparer l'avenir, et c'est bien regrettable ! La parole

Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, ce projet de loi de finances rectificative pour 2018 est bien une innovation attendue et positive dans notre procédure budgétaire. La nécessaire remise en ordre des comptes publics passe aussi par des adaptations des manières d'élaborer, d'autoriser, d'évaluer les textes budgétaires. Le sujet est sans doute moins médiatique que d'autres, mais il atteste en tout cas de la volonté du Gouvernement de transformer le pays et de financer chaque politique publique. Les collectifs de fin d'année n'étaient pas des jardins à la française, c'est le moins que l'on puisse dire ! Alors que ces textes étaient censés s'intéresser exclusivement à l'exercice en cours, des dispositions fiscales ne manquaient pas d'y fleurir, du fait tant des gouvernements, qui saisissaient souvent une occasion de rattrapage, que des parlementaires eux-mêmes, qui faisaient parfois un baroud d'honneur. Cela explique l'inflation du nombre d'articles dans les textes de ce genre : 96

il n'était pas rare que, du fait de la faiblesse des crédits votés en loi de finances initiale, les collectifs budgétaires soient assortis, pour répondre aux dépenses urgentes de l'État, de décrets d'avance qui, juridiquement, imposaient un vote de la représentation nationale. Pour la première fois depuis 1985, le Gouvernement a décidé de rompre avec ces pratiques : le texte ne comporte ni mesures fiscales ni décrets d'avance, ce qui a une portée politique particulière, avant la reprise sereine des débats sur nos institutions l'an prochain.

respect envers le Parlement, saisi de l'intégralité des ouvertures et des annulations de crédits budgétaires soumises à son autorité. Au Sénat, ce texte intervient en amont du projet de loi de finances pour 2019, sa discussion. Cet ordre met en évidence la cohérence de la trajectoire. Le texte n'a pas été adopté en commission, cela a été dit, et je le regrette, car à mon sens, vous vous en doutez, ce vote ne se justifie pas : des dépenses publiques constatées conformes aux prévisions, des évaluations de recettes fiscales et non fiscales sincères, des hypothèses macroéconomiques réalistes, autant d'ingrédients qui permettent aujourd'hui d'afficher une réduction du déficit public. Cette réduction est visible en valeur absolue, avec une prévision de déficit public de 80 milliards d'euros, contre 81,3 milliards d'euros prévus, et en valeur relative, ce qui correspond à un déficit de moins de 6 points de PIB pour 2018, alors que la trajectoire pluriannuelle la fixait à moins 2,8

de sécurité sociale, l'ACOSS, les intentions de recrutements en CDI ont augmenté de 10 % par rapport à l'an dernier, ce qui est une nouvelle bienvenue dans notre pays. Cela va aussi avec la réduction des cotisations sociales et le dégrèvement de la taxe d'habitation. L'impatience, voire la colère, on le voit, subsiste néanmoins. Le Président de la République l'a d'ailleurs reconnu. La France a trop tardé à réaliser ces transformations. Nous avons, me semble-t-il, souffert d'un attachement à une forme de « finances magiques » dans toute une série de politiques publiques. Ces travers ne sont pas totalement dissipés quand certains proposent ainsi la gratuité des transports publics, au hasard, sans dire combien ou comment ! Vous le savez bien, monsieur le ministre, si la solidarité est un objectif partagé, ce qui est le cas dans ce collectif à travers des ouvertures de crédits en faveur de l'hébergement d'urgence ou le soutien à la prime d'activité, elle doit être financée. Plutôt que la fuite en avant financière, nous préférons la transformation de l'action publique. Le Premier ministre a annoncé, le 29 octobre dernier, une stratégie ambitieuse pour les services publics, le fonctionnement et l'organisation de l'État sur la période 2018-2022. Je me félicite que chaque ministère se dote d'un plan de transformation numérique pour offrir une dématérialisation totale des démarches à l'horizon de 2022. L'objectif est de simplifier la vie de nos concitoyens, que ce soit avec la numérisation des ordonnances, la délivrance de baux numériques, la création facilitée des entreprises, tout en permettant des gains d'efficience pour la collectivité. Je trouve extrêmement positif que l'État se lance dans cette démarche à grande échelle, avec un portage politique au plus haut niveau. Il y a des expériences inspirantes à observer ; je pense notamment à l'Estonie, où les pouvoirs publics se sont engagés dans une stratégie numérique des services publics depuis quinze ans. L'Hexagone aime les silos. Je crois que nos concitoyens, notamment ceux qui sont nés après l'an 2000, sont attachés à l'agilité offerte par le numérique. L'idée n'est pas de reproduire des guichets sur la toile avec autant de mots de passe et d'interfaces ; il s'agit de plaider pour une « expérience utilisateurs » plus adaptée. Allégeons les démarches, facilitons la vie de nos concitoyens, changeons non les citoyens eux-mêmes, mais les procédures ! Ces initiatives ont déjà été amorcées dans la loi sur le droit à l'erreur. Au total, ce collectif budgétaire de fin d'année est l'occasion de rappeler une vérité : il n'est pas interdit de faire simple et de renoncer à de mauvaises pratiques. Comme l'écrivait Jean Cocteau : « Il n'y a pas de précurseur, il n'y a que des retardataires ». Bravo ! La parole

En effet, l'année dernière, je me suis engagé devant vous à ne pas prendre de décret d'avances- ce sera désormais la norme -et à ne prévoir aucune mesure fiscale dans le ce qui n'était jamais arrivé depuis l'adoption de la loi organique relative aux lois de finances, la LOLF. Nous voulons soumettre à l'approbation du Parlement des enveloppes budgétaires sincères, respectueuses des crédits inscrits en loi de finances que vous avez votés. Cette démonstration d'autosatisfaction devant l'effort accompli ne doit cependant pas faire oublier à tout un chacun qu'elle s'appuie sur un déficit public de 80 milliards d'euros, en hausse de près de 13 milliards d'euros par rapport à l'exercice précédent,

Plutôt que de s'interroger sur la progression du déficit de l'État, que l'amélioration- à quel prix ! -de la situation des comptes sociaux et de ceux des collectivités locales permet de masquer en grande partie, le Gouvernement préfère acter ses choix et se féliciter d'avoir réduit d'environ 6 milliards d'euros la prévision de déficit inscrite en loi de finances initiale. Le brevet de sincérité budgétaire que vous vous adressez est donc, de notre point de vue, largement écorné par celui de creusement des déficits et de la dette, que l'on doit également vous décerner. Le maintien de la contribution additionnelle de l'impôt sur les sociétés, sollicitée dans le collectif budgétaire du 1 décembre 2017, celui de l'impôt de solidarité sur la fortune et l'abandon du prélèvement libératoire forfaitaire sur les revenus du patrimoine auraient pu, ensemble, assurer au budget 2018 de se retrouver avec un point d'équilibre proche de celui du budget 2017. Autant de décisions anciennes pointées parmi les « gilets jaunes » ces jours-ci il y a belle lurette que, à l'instar d'autres qui vous ont précédé, vous avez choisi de mener à l'encontre de l'impôt une guerre d'attrition, l'éloignant toujours plus du lieu naturel de sa création- l'entreprise -pour investir largement les poches des consommateurs salariés ou retraités, sous forme de taxes à la consommation et de droits indirects,

Peut-être avez-vous aussi décidé de laisser à la loi de règlement le bonheur de revenir sur la réalité des chiffres, une fois passée la discussion d'un collectif toujours fixé sur une prévision de croissance qui ne va peut-être pas se réaliser. Revenons à l'essentiel. Le brevet de sincérité que vous vous êtes décerné ne peut masquer la nécessité d'ouvrir un certain volume de crédits supplémentaires, dans des domaines bien précis- je pense à la solidarité, à l'insertion, à l'égalité des chances, à la cohésion des territoires, à l'enseignement scolaire, au travail et à l'emploi où les urgences sociales semblent, encore une fois, avoir été insuffisamment évaluées en loi de finances initiale. Il ne peut pas davantage masquer le fait que certaines recettes fiscales ont connu une nouvelle baisse, notamment l'impôt sur les sociétés, les droits de mutation à titre gratuit ou encore l'impôt sur la propriété immobilière, ce croupion de l'ISF bien moins juste. Il a fallu la cession partielle des actions de l'État dans Safran, à hauteur de 1,2 milliard d'euros, pour que le compte final reste sur la crête des 80 milliards Ce mauvais choix pour l'industrie française, en motorisation aérienne comme pour l'électronique embarquée, est à ajouter à ce passif. Nous devrions être convaincus depuis bien longtemps que l'amélioration des comptes publics ne fait pas bon ménage avec ce portrait d'une France qui souffre de la précarité du travail, démultipliée par la réforme du code du travail, du mal-logement, produit d'une logique d'aide à la promotion immobilière et du véritable coup de bambou fiscal qui affecte l'ensemble de la fiscalité indirecte. Votre discours sur le pouvoir d'achat ne passe pas ! Il ne passe plus, ces temps-ci ! Nous ne voterons évidemment pas ce collectif, qui est, à nos yeux, un simple exercice d'autosatisfaction du Gouvernement. La parole est à M. Jean-Marc Gabouty.

de loi de finances rectificative allégé et recentré ne fait qu'ajuster l'équilibre de la loi de finances initiale par rapport à la prévision d'exécution. Contenant des dispositions d'ordre uniquement budgétaire, il met à jour les prévisions macroéconomiques pour l'année en cours, procède à des ajustements de recettes, certains comptes d'affectation spéciale et prévoit des ouvertures et annulations de crédits dans différentes missions. Jusqu'à présent, les lois de finances rectificatives servaient trop souvent d'exercice de rattrapage du budget de l'année, puisqu'elles contenaient de très nombreuses dispositions fiscales, sans impact effectif sur l'exercice budgétaire en cours. Les sous-budgétisations récurrentes lors des exercices précédents rendaient en effet nécessaire le recours aux décrets d'avance pour couvrir des dépenses urgentes. Le Gouvernement y a procédé une dernière fois au début de l'été 2017, et ce non-recours aux décrets d'avance en 2018 ne s'était pas produit depuis plus de trente valide donc les hypothèses macroéconomiques de la loi de finances initiale. Il s'appuie sur une prévision de croissance de 1,7 % du PIB, hypothèse, comme M. le rapporteur général légèrement optimiste. Certains organismes tablent en effet plutôt sur une croissance limitée à 1,6 %, avec une part acquise de 1,3 % à la fin du premier semestre 2018 2018 et un risque de tassement à l'automne, donc au dernier trimestre, particulièrement dans le secteur industriel. Quant à l'inflation, elle devrait, selon l'INSEE, s'établir à 1,9 % du fait, notamment, de la hausse du cours du baril de pétrole.

Les recettes budgétaires sont principalement améliorées par un supplément de recettes de TVA, ainsi que par une amélioration du produit des droits de succession et de donation pour partie imputable à une régularisation de comptabilisation de celles de l'exercice 2017, ce qui aurait dû donner un résultat un peu plus positif en 2017 et sans doute légèrement moins élevé cette année. En ce qui concerne les dépenses, malgré l'augmentation de celles-ci provenant de dépenses de personnel supplémentaires de certains ministères- 300 millions d'euros, ce qui n'est peut-être pas un très bon signe -, des montants plus élevés de la prime d'activité ou encore de dépenses d'urgence comme les surcoûts des opérations militaires, la réduction de l'objectif global de dépenses s'élèverait à 600 millions d'euros. On peut émettre des réserves sur certaines affectations ou sur un effort encore insuffisant de la réduction de la dépense publique, mais on ne peut conclure qu'à une exécution assez rigoureuse de la loi de finances initiale, ce qui est bien le rôle du projet de loi de finances rectificative. Pour ma part, je me félicite, en tant que rapporteur du compte d'affectation spéciale

En résumé, on ne peut être que satisfait, sur la forme, de la présentation de ce projet de loi de finances rectificative et, sur le fond, du résultat, qui se traduit par une réduction de 5,7 milliards d'euros du déficit budgétaire par rapport à la loi de finances initiale. Même s'il convient de relativiser ce chiffre au regard d'un déficit de 80 milliards d'euros, qui représente encore plus de 20 % de nos dépenses budgétaires, nous nous engageons quand même sur une trajectoire positive de la réduction des déficits. En conclusion, ce projet de loi de finances rectificative traduit une gestion plus saine et plus transparente, conforme aux engagements du Gouvernement et qui mériterait ainsi notre approbation.

une réalité qui ne surprendra que les amnésiques ayant oublié cette devise, sinon républicaine, en tout cas chiraquienne, qui pourrait être gravée sur le fronton de chaque ministère, au moins celui de l'économie et des finances

dans la fiscalité tentaculaire et confiscatoire, dans le creusement de la dette, sans même assurer ses fonctions régaliennes de défense extérieure et de sécurité intérieure, préférant augmenter les budgets destinés aux autres, plutôt que de répondre aux attentes légitimes et déjà anciennes des nôtres. Depuis samedi, nos compatriotes manifestent leur ras-le-bol d'être rackettés et, à l'image des élus locaux, ils demandent que vous cessiez, monsieur le ministre, de les prendre pour des imbéciles ! Comment ! Comment pouvez-vous faire preuve d'autant de cynisme, lorsque vous déclarez que les collectivités locales peuvent, si elles le veulent, baisser leur fiscalité, alors que vous n'avez eu de cesse, mais vous n'êtes pas le premier, de réduire la dotation financière de l'État aux communes, ce qui les conduit aujourd'hui à être fiscalement exsangues ? Dans ce contexte fiscal, il est impossible de relancer l'emploi- preuve en est le chômage, qui est officiellement reparti à la hausse. Pour le Gouvernement, les Français doivent faire des efforts, mais ils sont à bout de force, alors que la dépense publique, elle, n'a jamais été aussi élevée que cette année. Malgré tout cet argent pris dans la poche des Français, on taille dans le budget des armées, que l'on ampute de 400 millions d'euros ! La défense est priée de se charger seule de la totalité du coût des opérations extérieures et de Sentinelle, qui devait être initialement réparti entre tous les ministères. Et ce n'est pas une interview à bord d'un porte-avions qui changera quoi que ce soit à cette réalité financière et politique, qui freine encore et toujours la modernisation de nos troupes et met en péril ses capacités de défense du territoire national et de défense de nos intérêts à l'étranger. Cependant que l'on met les uns- toujours les mêmes ! -en coupe réglée, on trouve toujours de quoi alimenter la politique d'immigration dont nos compatriotes ne veulent pourtant plus : plus 11 millions d'euros au budget de l'Aide médicale de l'État, une AME en constante augmentation ; plus 80 millions d'euros pour financer l'aide aux demandeurs d'asile. Autant de financements qui auraient pu, qui auraient dû être attribués à l'équipement de nos soldats, mais que le Gouvernement préfère destiner à l'accueil de l'« Autre »- « l'Autre », encore et toujours ! Au vu de l'actualité marseillaise, qui peut encore oser affirmer que tout va mieux, mis à part quelques adeptes du gourou élyséen ? Du Havre à la cité phocéenne, communes fiscalement sinistrées, toutes deux à l'image de nombreuses collectivités mal gérées et surendettées, qui peut contester que nombre de nos territoires glissent vers un appauvrissement et un ensauvagement ? Dans le contexte national et international, qui peut dire que nous n'avons pas besoin d'une armée modernisée et de soldats parfaitement équipés ? Cet ajustement budgétaire de l'année en cours, mes chers collègues, nous donne à voir la réalité d'un quinquennat de continuité, sans aucune volonté d'opérer les changements majeurs que demande d'urgence la situation économique, sociale, sécuritaire

concrètement ? Eh bien, que l'intégralité des ouvertures et des annulations du schéma budgétaire pour 2018 aura été décidée par le Parlement. Nous renouons avec l'esprit de la LOLF, en respectant à la lettre le rôle central confié au Parlement en matière budgétaire : autoriser, contrôler et, de manière plus étroite encore, déterminer les dépenses. Ainsi, le rôle dévolu au Parlement est respecté, ce que nous tenons à souligner.

Nous tenons, avec l'ensemble des membres du groupe de l'Union Centriste, à saluer cette nouvelle donne. Elle est utile à la sincérité du budget, à la clarté de nos débats et à la lisibilité de la politique budgétaire de notre pays. Ce débat sur le chaînage vertueux des finances publiques et, de façon plus générale, sur l'agencement du calendrier budgétaire, nous aurons très certainement l'occasion de le prolonger lorsque seront examinés devant la Haute Assemblée les projets de loi constitutionnelle et organique. J'en viens 1,7 milliard d'euros d'ouvertures de crédits portant sur seize missions sur sept font l'objet d'une ouverture supérieure à 100 millions d'euros. Parmi celles-ci, l'indispensable ouverture de crédits, à hauteur de 150 millions d'euros, dans la mission « Cohésion des territoires »,

En revanche, comme l'a très justement relevé le rapporteur général de la commission des finances, nous nous interrogeons sur le rabot à hauteur de 577 millions d'euros des crédits alloués au compte d'affectation spéciale « Transition énergétique et ce, dans un contexte que nous connaissons et sur lequel je ne reviendrai pas, car nous aborderons le sujet lors de l'examen du projet de loi de finances initiale pour 2019.

L'objectif d'un déficit public à 2,6 points du PIB, c'est-à-dire en deçà du seuil fatidique des 3 %, est confirmé. Les prévisions initiales de croissance à 1,7 à 1,7 % sont également maintenues ; nous espérons bien entendu que ce taux pourra être atteint. Le niveau des dépenses pilotables de l'État est réduit à hauteur de 600 millions d'euros, ce dont nous nous réjouissons.

de l'article 11 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, qui a été inséré sur l'initiative de la commission des finances du Sénat. Cette disposition procède de la même logique redonner toute sa portée à l'autorisation et au contrôle parlementaires. En remettant en cohérence les plafonds d'emplois et les crédits de masse salariale votés en loi de finances initiale, elle en améliore la sincérité et l'effectivité. Dès l'année 2018,

Toutefois, à titre personnel, comme d'autres collègues de mon groupe, je voterai ce texte. En effet, nous tenons à insister sur l'effort de sincérité, donc de crédibilité, accompli par le Gouvernement dans la conduite de l'exercice budgétaire 2018.

Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, pour la première fois depuis trente ans, nous examinons un « vrai » projet de loi de finances rectificative. C'était un engagement du Gouvernement ; il a été tenu, et je m'en félicite. Jusqu'à cette année, les collectifs budgétaires de fin de gestion contenaient habituellement un grand nombre de dispositions fiscales nouvelles. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, et notre groupe n'a pas souhaité déroger à cette bonne pratique, qui fera, je l'espère, jurisprudence. De même, le Gouvernement n'a pas eu recours à des décrets d'avance. C'est une bonne décision, qui évite le mélange des genres entre projet de loi de

également la parole du chef des armées, qui avait pris des engagements très clairs vis-à-vis des armées durant la campagne présidentielle et lors des voeux aux armées. Cela reporte des programmes d'équipements indispensables à la sécurité de nos soldats et à l'avance technologique de nos armées. Certes, monsieur le ministre, j'entends bien l'argument de la nécessaire sincérisation du budget de la défense. J'entends aussi l'argument d'une hausse sans précédent du budget de la défense depuis de nombreuses années. J'entends encore l'argument du « dégel » récent de 272 millions d'euros de crédits de paiement pour le budget des armées, qui constitue un moindre mal.

Pour ce qui est des grands équilibres macroéconomiques, cela a été dit, la prévision de déficit public pour 2018 reste conforme à celle de la loi de finances initiale, soit 2,6 % du PIB. Néanmoins, l'effort structurel, lui, est pratiquement nul. C'est pourtant l'indicateur le plus pertinent pour mesurer l'effort de maîtrise des finances publiques. Nous aurons l'occasion d'avoir ce débat lors de l'examen du projet de loi de Nous souhaitons sincèrement que le processus Action publique 2022 que le Gouvernement a mis en place porte ses fruits. Nous souhaitons sincèrement que l'objectif de 50 000 fonctionnaires en moins d'ici à la fin du quinquennat soit tenu. Nous souhaitons sincèrement que le combat pour l'assainissement des comptes publics soit mené à bien,

Les Français demandent de la clarté et de la pédagogie. Ils demandent surtout des réformes supportables, utiles et qui leur paraissent acceptables. Changer de modèle est toujours difficile, monsieur le ministre. C'est même une mission historique pour votre gouvernement. Les choix doivent être faits de façon pragmatique, en tenant compte de la réalité et du quotidien des Français. Nous espérons donc que vous entendrez ces derniers. Sous réserve de l'adoption de notre amendement relatif à la mission « Défense », je ne vois pas de raison de s'opposer

la décision du Gouvernement de faire supporter le surcoût des OPEX par le budget de la défense, et non pas, comme la loi le prévoit, par la solidarité interministérielle.

un courrier personnel de M. le Premier ministre. J'y ai été évidemment particulièrement sensible, même si, vous le comprenez, monsieur le ministre, nous ne pouvons partager les éléments contenus dans cette lettre. Je veux saluer ici aussi les efforts constants de Mme la ministre des armées, qui, depuis sa prise de fonction, a marqué sa ferme volonté de redonner à nos armées leurs capacités opérationnelles depuis trop longtemps défaillantes. Nous nous sommes engagés à ses côtés. Certes, l'exercice budgétaire 2018 se termine dans des conditions meilleures que l'an passé pour le budget des armées, mais, compte tenu de l'immensité des besoins à couvrir, on ne peut pas se satisfaire de cette situation

ministre, vous avez multiplié les explications pour tenter de nous rassurer et nous expliquer que la disparition de 404 millions d'euros n'avait aucun impact sur les engagements du Gouvernement pour la remise à niveau de nos armées. Vous déclarez : « La loi de finances pour 2018 sera exécutée à l'euro près ».

qui seront soit reportées, soit annulées. On savait dès le début que l'enveloppe réservée aux OPEX était insuffisante ; le Sénat l'avait dit ! Aujourd'hui, on demande aux armées de payer les opérations Barkhane- 700 millions d'euros -, Chammal- 460 millions d'euros -et Sentinelle- 215 millions d'euros -, avec des dépenses initialement prévues pour la modernisation de l'équipement, la réparation d'infrastructures vétustes ou l'amélioration de la condition de vie en régiment. Le nier est inutilement blessant pour nos armées, qui peuvent comprendre que l'on perde un arbitrage budgétaire, mais pas que l'on déguise la vérité. Vous déclarez par ailleurs, monsieur le ministre : « En 2019, le budget sera conforme à la première annuité de la LPM ». Un enfant d'école primaire comprendrait que des dépenses reportées de 2018 à 2019 réduiront d'autant l'augmentation réelle des moyens ! Nos débats pendant l'examen de la LPM ont montré les immenses besoins d'un outil militaire fatigué, quand il n'était pas à bout de souffle, à force de suremploi et de sous-investissement. Ainsi, pour les seules infrastructures, l'état des casernes par exemple, les besoins non couverts sur la programmation sont chiffrés par notre commission à 1,5 milliard d'euros. l'on ne nous dise pas qu'il y avait de la marge. C'est faux ! Le Gouvernement tend à nous expliquer qu'il n'y aura pas de conséquences physiques, voire que le ministère des armées serait satisfait que l'on lui prenne 400 millions d'euros : voilà qui laisse évidemment bouche bée ! Dans ce cas, si le Secrétariat général pour l'administration n'arrive pas à dépenser ces crédits, qu'il laisse donc la main aux commandants des bases de défense, qui sont parfois obligés de remonter à Paris pour faire face à des réparations d'infrastructures, de bâtiments, de cantine ou de transport automobile de leurs soldats. Quant aux difficultés de recrutement, comment ne pas voir qu'elles résultent de la faible attractivité de carrières où l'engagement est total, mais la rémunération insuffisante ? Les médecins militaires quittent le service militaire aux armées pour augmenter leur rémunération. Des réformes s'imposent ; nous attendons du Gouvernement des annonces en ce sens.

En conclusion, la légèreté avec laquelle le Gouvernement a rayé d'un trait de plume 404 millions d'euros de crédits a quelque peu ébranlé notre confiance. Plus grave encore est l'impact politique que cette décision risque d'avoir.

Tout cela augure bien mal de l'avenir. Le Sénat a accompagné les efforts de Mme la ministre des armées, pour que, enfin, la sincérité de nos engagements soit synonyme de vérité.

comme le Gouvernement s'y était engagé, ce collectif de fin de gestion ne comprend pas de dispositions fiscales nouvelles. C'est un progrès sensible par rapport aux années précédentes,

se limite à neuf articles et, pour l'essentiel, à de simples mesures budgétaires ajustant l'équilibre de la loi de finances initiale. Si le délai d'analyse reste court, ... C'est vrai. ... il est cependant aujourd'hui plus conforme à la nature même du texte. J'en viens au scénario macroéconomique. Le Gouvernement conserve sa prévision de croissance à 1,7 %, peut-être légèrement optimiste, mais le risque n'est sans doute pas significatif sur le plan budgétaire.

Si le solde budgétaire connaît par ailleurs une légère amélioration, il le doit pour l'essentiel à la vente de 2,35 % du capital de Safran et à l'accroissement des recettes perçues par l'État au titre de la taxe intérieure de consommation sur les Opération ponctuelle pour l'une, recette de constatation pour l'autre : rien ne justifie que le Gouvernement ne se félicite pas particulièrement de cette amélioration du solde budgétaire.

spéciale « Transition énergétique », s'il n'y a pas lieu de s'offusquer du rééquilibrage budgétaire opéré, il convient cependant de s'étonner d'une sous-consommation des crédits à hauteur de 600 millions d'euros, donc de la réversion d'une part de TICPE au budget général, au moment où chacun s'interroge sur les montants de fiscalité écologique prélevés au regard des actions menées en matière de transition énergétique. Nous déposerons donc un amendement- d'appel, bien évidemment -pour évoquer ce sujet avec vous, monsieur le ministre. Ma collègue Hélène Conway-Mouret vous interrogera sur le budget de la mission « Défense ». Pour ma part, permettez-moi seulement de m'étonner que la prise en charge des OPEX et de l'opération Sentinelle se fasse essentiellement par annulation de crédits, notamment ceux qui sont dédiés à l'équipement des forces, dont je pensais qu'ils avaient été sanctuarisés. Mais oui ! C'est en tout cas la lecture que j'avais faite de la toute récente loi de programmation militaire.

Pour ce qui concerne la mission « Travail et emploi », la baisse très significative des crédits de la mission pour 2019 se double d'une annulation de crédits de paiement pour 2018 de près de 500 millions d'euros. La justification de ces annulations de crédits reposerait sur l'amélioration de la conjoncture. Nous nous en réjouirions avec vous, monsieur le ministre, si tel était bien le cas. Or plusieurs amendements de rétablissement des crédits de la mission nous permettront de démontrer qu'il n'en est rien. Ainsi, 359 millions d'euros sont annulés pour le programme 102, qui concerne les contrats aidés et l'insertion par l'activité économique. Au total, la baisse réelle de ce programme aura été de 953 millions d'euros en crédits de paiement par rapport à 2017. Rappelons-nous que la loi de finances 200 000 contrats aidés en 2018, en diminution de 100 000 par rapport à 2017, avec, qui plus est, un taux moyen de prise en charge par l'État de 50 % du SMIC brut en 2018, contre 72 % en 2017. Comment d'ailleurs s'étonner que, dans ces conditions, des crédits n'aient pas été utilisés, supprimant des occasions d'entrer dans le monde du travail pour les publics concernés et mettant en difficulté des secteurs associatifs liés à la culture, à la petite enfance ou aux soins à domicile par exemple ? En pratiquant en deux fois, le Gouvernement a voulu masquer l'importance de la baisse réelle concernant les contrats aidés. Il a, de fait, caché ses intentions réelles au Parlement. Sincérité budgétaire, disiez-vous, monsieur le ministre L'annulation des crédits mis en réserve pour l'aide à l'embauche dans les PME sera aussi pour nous l'occasion de vous interroger sur la suppression d'une mesure qui aurait sans doute mérité d'être ajustée en étant ciblée davantage vers les toutes petites entreprises, afin d'en limiter les effets d'aubaine.

Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, affecte principalement en annulations de crédit deux missions : « Travail et emploi » et « Défense ». Sur la première mission, à l'évidence, il s'agit d'une sous-exécution des dispositifs d'aide à l'emploi, qui pose de nouveau la question de leur efficacité.

Certes, la provision OPEX était majorée de 200 millions d'euros en 2018 par rapport à 2017, mais la solidarité interministérielle qui prévalait par le passé, si elle n'exonérait pas les armées de participer au financement des OPEX, en limitait le coût-

Si je considère la sous-consommation des crédits de personnels pour 150 millions d'euros, sujet sur lequel nous aurons l'occasion de revenir, car il témoigne d'un double phénomène- difficultés à recruter et à fidéliser les personnels -, ce sont encore 430 millions d'euros d'amputation, soit le record des sept dernières années.

un spécialiste de la comptabilité publique. Moi non plus ! Je compte peut-être comme un épicier breton, ne m'en voulez pas ! Mais je ne vois pas comment, en annulant des crédits de paiement, nous pourrons honorer en temps et heure nos factures. De la même façon, je ne vois pas comment l'annulation d'autorisations d'engagement ne se traduira pas à un moment ou à un autre, en 2019, 2020 ou 2021, par des retards dans les livraisons. En conclusion, si ce bonneteau touchait d'autres missions que la mission « Défense », je n'y verrais qu'une technique budgétaire peu glorieuse pour boucler le budget. Le problème, c'est que nous touchons à la défense, fonction régalienne par définition, fonction dont le Président de la République est le garant. Remonter les Champs-Élysées dans un command-car ou s'adresser aux Français depuis le fleuron de la marine française, c'est bien. Toutefois, on attend du chef suprême des armées non qu'il nous livre de belles images de lui en situation, mais qu'il respecte sa parole. Déclarer la main sur le coeur que l'on veut sanctuariser les crédits de la défense, inviter nos partenaires européens à construire une défense européenne nécessite de mettre en cohérence ses actes et ses paroles. C'est sa crédibilité de chef d'État et de chef des armées qui est en cause. Décidément, en matière de pratique budgétaire, le

Votre emploi abusif de superlatifs, monsieur le ministre, crée de grands espoirs et provoque une déception d'autant plus grande. Elle crée aussi, dans tous les domaines, un écran de fumée derrière lequel vous vous cachez pour mieux tout casser. Quand il se dissipe, on découvre trop souvent une autre réalité, différente de celle que vous avez annoncée.

Cette disposition qui primait jusqu'alors est pourtant inscrite en toutes lettres dans l'article 4 de la loi de programmation militaire, promulguée au mois de juillet dernier. C'est donc en toute bonne foi que nous avons voté ce texte et que nous avons voulu croire dans les promesses qui nous étaient faites, celles d'un effort inédit, d'une remontée en puissance exceptionnelle et d'un renouveau du budget des armées, éléments de langage certes utilisés par tous les ministères, mais qui semblaient appropriés au vu des chiffres annoncés. Il a donc suffi de quatre mois pour balayer cet engagement au détour d'un projet de loi de finances rectificative. Monsieur le ministre, vous justifiez ce revers par votre volonté de sincérisation et de responsabilisation budgétaire- en tout cas, ce sont les mots-clefs, à en juger par l'utilisation que vous en avez faite dans vos propos. J'entends, dans ce discours, une subtile hâblerie, autrement plus habile que les violentes coupes budgétaires à hauteur de 850 millions d'euros survenues à l'été 2017, qui avaient poussé à la démission le chef d'état-major des armées. Comment parler de sincérité quand le budget alloué aux OPEX est de 650 millions d'euros, alors que leur coût réel atteint 1,2 milliard d'euros ? été plus honnête d'annoncer une augmentation du budget des armées pour 2018, non de 1,2 milliard d'euros, mais de 800 millions d'euros. De même, est-ce responsabiliser un ministère que de l'affaiblir en lui coupant ses crédits ? ? Derrière ce que l'on nous présente froidement comme un simple exercice comptable, je vois l'impact direct de cette mesure sur nos militaires. Alors que nous leur certifiions hier la préservation de leurs moyens, ils devront aujourd'hui composer avec une baisse de 319 millions d'euros alloués à l'équipement des forces, avec un inévitable report des commandes. Nous connaissons leurs besoins en matériel pour assurer leur sécurité et la nôtre, mais ils devront encore attendre. Je regrette que l'engagement que nous avons pris collectivement avec la LPM au mois de juillet dernier soit foulé aux pieds, que le vote du Parlement soit rendu caduc et, surtout,

on a envie de remettre au Gouvernement une médaille ... Oui, la médaille du respect de l'écoute du Parlement. Dans une médaille, il y a l'avers et le revers.

prochaine. La discussion générale est close. J'informe le Sénat qu'une candidature pour siéger au sein de la commission des lois a été publiée. Cette candidature sera ratifiée si la présidence n'a pas reçu d'opposition dans le délai d'une heure prévu par notre règlement.

monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, le Haut Conseil des finances publiques pointe une forme de stagnation du résultat des efforts accomplis et demandés à la grande majorité de nos compatriotes. Il écrit : « Les recettes font l'objet d'ajustements à la hausse pour les droits de mutation à titre onéreux et pour les recettes non fiscales et à la baisse pour les droits de succession et de donation ainsi que pour l'impôt sur la fortune immobilière. Les recettes de TVA encaissées sur les neuf premiers mois de l'année sont en retrait par rapport à la prévision. « Un rattrapage important est attendu par le Gouvernement d'ici à la fin d'année, en lien notamment avec le rebond prévu de la consommation des ménages et un rythme moins élevé des remboursements et dégrèvements qu'à la fin 2017. Le Haut Conseil considère que l'ampleur de ce rattrapage pourrait être plus modérée. « La prévision des autres recettes est globalement en ligne avec les informations disponibles- encaissement des recettes fiscales, prévision de masse salariale de l'ACOSS, l'Agence centrale des

Une telle situation nous conduit, mes chers collègues, non à une conversion aux mérites du processus actuel d'analyse des documents budgétaires, mais à une conclusion simple. La priorité accordée par le Gouvernement à l'allégement des obligations fiscales des entreprises et des particuliers les plus fortunés ne semble pas s'être traduite en termes de croissance et d'investissements, ces derniers étant annoncés en stagnation cette année.

! Nous ne pouvons pas, de notre point de vue, améliorer durablement la situation des comptes publics si nous ne passons pas par une grande remise à plat de notre fiscalité, laquelle est nécessaire pour rétablir l'égalité et la justice fiscales, promouvoir l'efficacité économique et sociale de l'impôt et assurer son utilité.

pour l'initiative économique, les fonds d'investissement de proximité sont des véhicules qui doivent investir 70 % de leurs actifs pour renforcer les fonds propres ou quasi propres de PME non cotées, à tous les stades de leur développement. En 2007, le législateur, constatant qu'aucun des FIP levés en quatre ans n'avait choisi d'investir en Corse, a créé le FIP Corse. Ce véhicule devait, grâce à un dispositif fiscal plus avantageux que sur le reste du territoire français, orienter l'épargne des Français et mettre enfin la Corse sur les routes de la finance. Près de douze ans se sont écoulés, et nous pouvons, à la lumière des chiffres, considérer que ce dispositif s'est révélé fructueux, étant entendu que l'attractivité du FIP Corse repose sur son différentiel de vingt points par rapport aux FIP nationaux. Les montants collectés, une quinzaine de fonds gérés par cinq sociétés de gestion différentes, se montent aujourd'hui à près de 380 millions d'euros. On estime que les sociétés financées par les FIP Corse représentent 2 000 emplois directs en Corse, et même 7 000 si l'on y ajoute les emplois induits. Jusqu'en 2018, les taux de réduction étaient de 38 % pour la souscription d'un FIP Corse, contre 18 % pour un FIP finançant des entreprises continentales. Niveler cet avantage sur l'ensemble du territoire français reviendrait à refaire de la Corse un désert financier. Pour rester attractif, le FIP Corse doit nécessairement maintenir son différentiel de vingt points par rapport aux FIP nationaux.

doivent se concrétiser dans les prochaines semaines. Bruno Le Maire fait ce travail très important avec la Commission. La mesure prise par le Gouvernement n'est donc effectivement pas entrée en vigueur, pour la raison que vous évoquez très justement, monsieur le rapporteur général.

l'article. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, de deux choses l'une : ou bien les sommes consacrées à la transition énergétique procèdent de l'affichage parce que l'écologie est dans l'air du temps, ou bien, comme nous le pensons, la fiscalité à vocation écologique permet, sans difficulté majeure, de créer l'un de ces chapitres réservoirs dont notre droit fiscal est affublé. Prenons l'histoire récente du compte d'affectation spéciale « Transition énergétique », dont il est question à cet article 2.

En 2017, alors que la loi de finances initiale avait inscrit près de 40 % des recettes de la TICPE dans le périmètre des ressources du compte, la correction a atteint 862,3 millions d'euros en net, une partie de la réduction ayant finalement été mobilisée par EDF pour payer l'effacement des factures de certaines entreprises. En 2018, la correction atteindra 577,6 millions d'euros.

Si la fiscalité écologique dédiée se révèle surdimensionnée au regard des besoins, il faut la réduire. En tout cas, il faut cesser d'en faire une simple variable d'ajustement.

est à M. Claude Raynal. Il s'agit très clairement d'un amendement d'appel. Nous avons parfaitement conscience de l'inutilité de la constitution d'un surplus budgétaire au sein d'un compte d'affectation spéciale. L'article 2 prévoit un ajustement de la part de TICPE

Le Gouvernement justifie cette affectation de recettes par une décision de la Commission de régulation de l'énergie de juillet dernier, qui estime que les compensations de charges au titre de 2018 seront inférieures de 600 millions d'euros à ce qui était prévu. Sur le fond, nous estimons, compte tenu de l'urgence du défi écologique, qu'il est nécessaire que les recettes de la fiscalité écologique soient redirigées autant que possible vers des actions en faveur de l'environnement. Au lieu de réaffecter ce demi-milliard d'euros- ce n'est pas une petite somme ! -au budget général, n'aurait-il pas fallu accroître les politiques publiques en faveur de la transition écologique ?

un élargissement des critères de prise en charge financière, afin de soutenir les entrepreneurs dans leur démarche novatrice. C'est à l'État qu'il appartient parfois de prendre des risques en matière d'innovation. Pour tout vous dire, mes chers collègues, je préfère un État qui aide des entreprises audacieuses à un État qui consolide des rentes de situation dans des secteurs qui n'en ont nullement besoin, comme c'est quelquefois le cas

Quel est l'avis de la commission ? La commission comprend, bien évidemment, l'intention de Claude Raynal, qui a d'ailleurs très justement indiqué qu'il s'agit d'un amendement d'appel. Très concrètement, la Commission de régulation de l'énergie a considéré dès le mois de juillet

Si le Sénat n'adopte pas l'article d'équilibre, il ne pourra pas, sauf demande de seconde délibération portant sur cet article, voter en faveur de la première partie. En effet, en application de la loi organique relative aux lois de finances, et conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, la première partie doit avoir été adoptée « en celles de ses dispositions qui constituent sa raison d'être Il en est ainsi de l'article 4, qui arrête en recettes et en dépenses les données générales de l'équilibre. Il s'agit donc d'un vote de cohérence. En revanche,

le Sénat n'a pas adopté l'article d'équilibre. Puis-je considérer qu'il rejette en conséquence la première partie loi ? Le Sénat n'ayant pas adopté la première partie du projet de loi de finances rectificative pour 2018, l'ensemble du projet de loi est considéré comme rejeté.

Débat sur la diplomatie climatique de la France à l'aune de la COP24. Explications de vote puis vote des groupes sur la proposition de loi visant à lutter contre l'exposition précoce des enfants aux écrans,